est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2021. Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions.

et, malgré le désastre qu'a été l'année 2020 du fait de la crise sanitaire, ils sont plutôt satisfaits de la manière dont ils sont soutenus. Évidemment, madame la ministre, avec une petite réserve : ils comprennent bien, pour la plupart d'entre eux, vous pardonnerez l'anglicisme, que c'est une aide, une aide, et ils rêveraient d'une augmentation du budget plutôt que de crédits conséquents dans un plan de relance qui, par définition, ne devrait pas être reconduits l'année prochaine.

j'ai trouvé, madame la ministre, les responsables de ce centre extrêmement actifs, dynamiques, très portés sur le soutien au cinéma, mais aussi à l'industrie cinématographique, aux producteurs,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous me permettrez d'évoquer la situation financière des opérateurs de l'audiovisuel public extérieur. Si la crise sanitaire a pu avoir des effets paradoxalement positifs en 2020 sur les comptes de France Médias Monde (FMM), lui permettant, grâce à la diminution des dépenses et au report de certains projets, d'accélérer la reconstitution de ses capitaux, les perspectives à moyen terme demeurent incertaines. En effet, la baisse des ressources propres, liée à la crise économique, pourrait avoir des effets sur l'équilibre financier des opérateurs. D'ores et déjà, la chaîne TV5 Monde a été affectée en 2020 par la diminution de ses recettes publicitaires et des recettes de distribution liées à la vente de programmes. Dans ce contexte, la diminution, pour FMM, et la stagnation, pour TV5 Monde, des dotations prévues par le projet de loi de finances pour 2021, certes conformes à la trajectoire financière définie en 2018, ne sont évidemment pas une bonne nouvelle. L'évolution à la baisse depuis plusieurs années de leurs ressources publiques fragilise les sociétés de l'audiovisuel public extérieur, confrontées confrontées à une augmentation mécanique de certains de leurs coûts et à la concurrence internationale d'autres opérateurs. En 2020, a reçu une dotation de 373 millions d'euros, d'euros, et la une dotation de 362 millions d'euros, soit plus de 100 millions d'euros de plus que FMM ! Sans parler des soutiens que reçoivent les médias extérieurs des États puissances. Dans le même temps, les ambitions affichées ne sont pas revues à la baisse, comme en témoignent les nouveaux plans stratégiques des deux sociétés. Cette situation oblige les deux opérateurs à faire des choix difficiles,

De la même manière, TV5 Monde a dû réduire récemment sa couverture satellitaire en Europe orientale et en Asie centrale. Les performances accomplies par les opérateurs de l'audiovisuel public extérieur n'en restent pas moins méritoires. En 2019, FMM a vu le nombre de « contacts hebdomadaires » sur ses trois médias progresser de 18 %, la hausse frôlant les 38 % sur le segment numérique. 2019, la chaîne France 24 en espagnol est passée d'une diffusion de six heures à douze heures par jour à budget constant, permettant une hausse de moitié du nombre de téléspectateurs hebdomadaires. C'est une grande avancée, qui ancre France 24 en Amérique latine. Au final, je veux rendre hommage aux opérateurs de l'audiovisuel extérieur, qui, avec des moyens modestes, jouent un rôle important pour notre rayonnement. Nous devons impérativement les soutenir et les défendre sur le plan budgétaire.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite également insister sur la spécificité de la mission des opérateurs de l'audiovisuel public extérieur porter le rayonnement de la France ; d'autre part, promouvoir nos valeurs et notre langue dans le monde. Et c'est dans ce cadre que France Médias Monde intègre dans sa ligne éditoriale la thématique relevant de nos valeurs démocratiques et républicaines. Ainsi, après l'assassinat de Samuel Paty, l'opérateur a su bouleverser ses programmes et mettre en exergue les actions d'éducation aux médias et à l'information. Comment procède-t-il ? D'abord, par le développement de la diffusion en langues étrangères, notamment les langues africaines et la langue arabe. Ensuite, par le développement de la francophonie, axe politique fort partagé avec TV5 Monde. Et le tout s'accompagne d'une implication dans la lutte contre la désinformation. Il est dans l'ADN de nos opérateurs de défendre nos valeurs. Cet engagement intransigeant et déterminé les expose à de nombreuses menaces. Ils sont ainsi régulièrement la cible de cyberattaques. Souvenons-nous de celle qui a visé TV5 Monde en 2015. Elles sont désormais un phénomène durable et ancré. FMM a dû affronter jusqu'à 400 000 tentatives d'intrusion entre mai et juillet 2019, et profite depuis d'une certaine « stabilisation », avec seulement 300 000 tentatives par mois. Sur le terrain, personnels et correspondants sont des cibles privilégiées. Entre 2000 et 2013, quatre journalistes de Radio France internationale (RFI) ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et chaque année, on recense de multiples cas d'agressions, voire d'emprisonnements, à l'instar de la situation du journaliste algérien Khaled Drareni, correspondant de TV5 Monde, en prison depuis le mois de mars 2020. Malgré un niveau de dangerosité dans le monde qui ne faiblit pas, nos opérateurs sont déterminés à poursuivre leurs missions avec une ambition à hauteur des moyens qui leur seront alloués.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'année 2020 devait être celle de la « grande loi » audiovisuelle. Le temps semblait venu de mettre un terme aux désordres nés de l'absence de pilotage stratégique et de la multiplication des tutelles. Cette réforme de la gouvernance devait s'accompagner d'une réforme du financement, au travers de la modernisation de la contribution à l'audiovisuel public (CAP). Votre prédécesseur, madame la ministre, nous avait assuré voilà deux ans que la réforme de la CAP aurait lieu dans le PLF 2021 au plus tard À ce stade, une formule du génial Edgar Faure me vient à l'esprit pour qualifier la situation de l'audiovisuel public français : « Voilà que s'avance l'immobilisme, et nous ne savons comment l'arrêter. En revanche, nous savons aujourd'hui que le Gouvernement a renoncé à réformer efficacement le secteur de l'audiovisuel. Ce renoncement constitue d'abord un choix du Gouvernement, et non une conséquence de la crise sanitaire. Non seulement ces deux réformes auraient pu être engagées plus tôt dans le quinquennat, mais il restait encore suffisamment de temps pour les mettre en oeuvre d'ici à 2022. Le seul horizon de votre majorité semble donc être celui de la trajectoire budgétaire 2018-2022,

C'est évidemment insuffisant pour faire face à l'offensive des plateformes américaines, qui engrangent des millions d'abonnés et devraient prochainement accroître l'attractivité de leurs offres en programmes français.

Notre secteur des médias est en danger, et le Gouvernement semble détourner le regard en considérant qu'il n'y a pas d'urgence. Or la crise sanitaire est venue rappeler que la grande dépendance des sociétés de l'audiovisuel public au développement de leurs ressources propres pouvait constituer une véritable Un service public a besoin de stabilité et de prévisibilité pour développer ses missions ! Depuis 2017, c'est un surcroît de précarité qui leur a été proposé ! Une remise à plat des modèles économiques n'a jamais été aussi nécessaire. Nous étions prêts à ouvrir ce débat au Sénat. au Sénat. Par exemple, la suppression à terme de la publicité sur les antennes publiques pour la réserver aux chaînes privées conserve toute sa pertinence. Madame la ministre, nous ne partageons pas le manque d'ambition du Gouvernement pour l'audiovisuel public, et nous regrettons le temps perdu jusqu'à la fin du quinquennat. Ce désaccord stratégique n'est pas contradictoire avec quelques satisfecit. Nous soutenons ainsi l'enveloppe de 70 millions d'euros issue du plan de relance, ainsi que l'intention du Gouvernement de négocier avec les entreprises de l'audiovisuel public des contrats d'objectifs et de moyens (COM) sur la période 2020-2022 comportant enfin des objectifs communs. Si notre commission a considéré que le Gouvernement pouvait et devait mieux faire en matière d'audiovisuel, elle a toutefois émis, mais- vous l'aurez compris -sans entrain, un avis favorable à l'adoption des crédits du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » du projet de loi de finances pour 2021.

reviendrai donc pas sur l'analyse des crédits, excellemment réalisée par notre collègue de la commission des finances. Cependant, et je veux le souligner, la presse n'a pas été oubliée par la solidarité nationale, et les professionnels en ont pleinement conscience. Chaque acteur de la filière a ainsi exprimé, sinon sa pleine satisfaction, du moins sa reconnaissance de l'effort fourni. Je pense aux diffuseurs, aux vendeurs et aux éditeurs. J'ai choisi de mettre en avant trois points qui me paraissent essentiels premier concerne l'avenir de la distribution. L'année 2020 a vu la cessation d'activité, annoncée de longue date, de Presstalis. À l'heure actuelle, nous sommes encore incapables de chiffrer le coût global pour les finances publiques du soutien apporté ces dernières années à cette entreprise, mais il est probablement La responsabilité des éditeurs, qui ont géré la société, ne peut pas être écartée. Mais ils en paient aujourd'hui le prix fort avec, pour quasiment tous, des pertes liées aux créances de Presstalis. Preuve est faite, selon moi, des dangers d'un soutien public massif quand il n'est pas associé à une authentique réforme. À la fin, et en l'absence de vision partagée, cela a accru le déficit, pour un résultat médiocre. Dès lors, je suis encore inquiet sur l'avenir de la nouvelle société. Peut-on raisonnablement avoir sur un marché en attrition constante deux sociétés, France Messagerie et les Messageries lyonnaises de presse (MLP), d'autant plus que de nouveaux acteurs pourront s'y joindre dans les années à venir ? Cette interrogation reste largement ouverte. deuxième point porte sur les droits voisins des éditeurs et des agences de presse. Sur ce dossier, à l'origine duquel se trouve la proposition de loi de notre collègue David Assouline, les bonnes nouvelles succèdent aux reprises de procès, qui entraînent eux-mêmes une prolongation des négociations. Soyons clairs : il est impératif pour la France et pour l'Europe de faire respecter le droit. Il faut donc que cette législation soit appliquée, faute de quoi le dernier pan de notre souveraineté s'effondrera. Mais soyons aussi honnêtes : les droits voisins ne résoudront pas à eux seuls la crise profonde que traverse la presse, pas uniquement en France, cette crise étant amplifiée par la pandémie. Là encore, je compte rester vigilant, en lien avec les professionnels, pour garantir que la volonté des législateurs européen et national ne sera pas étouffée au détour d'un accord

Voilà, madame la ministre, une bonne façon de préparer un avenir où devront cohabiter une presse papier, que l'on espère stabilisée, et une presse numérique, qui a accéléré son développement à la faveur du confinement, mais qui doit encore travailler à son

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, au début de l'année 2020, il aurait fallu un scénariste particulièrement inventif pour imaginer le scénario catastrophe de la pandémie avec laquelle nous vivons. Comme tous les secteurs de l'économie, la crise frappe le monde du cinéma dans son ensemble. Elle sape ce plaisir simple de profiter, seul ou entre amis, d'un bon film. La France a présidé à la naissance du grand écran, entre La Ciotat des frères Lumière et la fondation du groupe Pathé la même année à Vincennes, ville chère au coeur de notre président de commission. Il faut ainsi rappeler le lien très fort qui nous unit à notre cinéma. En Europe, notre pays est de loin celui qui accueille le plus de spectateurs et où la part de la production nationale est la plus importante. C'est dire que la préservation de notre modèle est essentielle,

Il a permis à la production française de ne pas s'interrompre totalement. Ensuite, des mesures ont été prises en faveur des salles de cinéma. Je note cependant que les cinémas municipaux n'ont qu'un accès très réduit, « au cas par cas », à ce fonds de compensation,

des négociations actuellement menées autour de la transposition de la directive SMA, qui doit à tout prix réserver une place au cinéma, peut-être au travers d'une nouvelle chronologie des médias conciliant les intérêts des grands acteurs historiques de notre création et ceux des nouveaux entrants.

Comme souvent, il y a les mots, les mots, et puis ... Et puis, il y a le budget ! Il y a les éloges pour le service public de l'audiovisuel, pour ses missions essentielles pour la citoyenneté et les valeurs de la République, pour l'exigence et la diversité culturelle, pour son rôle éducatif

non seulement à cette crise, qui- nous l'espérons -est conjoncturelle, mais à une concurrence qui est non plus uniquement celle du privé, mais celle de géants du net. À eux seuls, ces derniers ont la puissance financière d'États et de nations riches. Je le dis franchement, vous avez abandonné toute ambition pour le service public de l'audiovisuel, pas seulement en réduisant son budget, alors que les recettes publicitaires manquent à cause de la pandémie, mais en abandonnant dans le même temps la grande réforme annoncée de l'audiovisuel et celle de la redevance, une redevance que vous continuez en plus à baisser par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Vous le faites alors que les États européens qui nous entourent non seulement ont réformé la redevance, devenue ainsi universelle, mais perçoivent un montant nettement supérieur au nôtre plus 180 euros au Danemark, plus 78 euros en Allemagne, plus 38 euros au Royaume-Uni, quand vous mégotez pour un ou deux euros qui rapporteraient 30 à 60 millions d'euros supplémentaires directement affectés au financement de notre audiovisuel public. C'est ainsi que vous remerciez les résultats d'audience remarquables et la qualité des programmes de plus en plus remarquée de Radio France et France Télévisions, qui ont réalisé pourtant tant de sacrifices, d'efforts et d'économies depuis plus de cinq ans. Ces baisses ne sont pas nouvelles. C'est une trajectoire budgétaire que votre gouvernement a imposée depuis plusieurs années et que vous allez poursuivre froidement, y compris dans les circonstances dramatiques d'aujourd'hui. Vous proposez que l'audiovisuel public connaisse une perte de 69 millions pour 2021 alors que sa dotation était déjà en baisse de 3,36 % en 2020. Avec une telle trajectoire, même le niveau d'investissement dans la création, qui était jusqu'à maintenant préservé, ne pourra plus l'être demain. Déjà, les émissions de flux, d'information et de sport, qui consacrent pourtant plus que jamais la télévision en linéaire, sont rognées. Après la fermeture de France Ô et celle, programmée, de France 4, vous continuez à affaiblir dans les faits notre audiovisuel public. C'est la réalité ! Avec des amis comme ce gouvernement, l'audiovisuel public n'a pas besoin d'ennemis. Je veux maintenant aborder l'aide au cinéma, qui continuait à enregistrer de bons résultats avant la crise sanitaire, avec une croissance de 18 % à l'export en un an, et le deuxième plus haut niveau de fréquentation des cinémas depuis cinquante-trois ans en 2019, avec 213,3 millions d'entrées. Mais, en 2020, sous les effets de la pandémie elle-même et des mesures sanitaires chaotiques qui ont été imposées, le cinéma vit une situation dramatique, avec une baisse de plus de 50 % des fréquentations des salles, le tout entraînant notamment des reports de film.

Je salue les aides du plan de relance et la progression non négligeable de 11,6 millions d'euros des crédits liés au programme « Livre et industries culturelles ». Je vous demande tout de même- c'est l'objet de deux amendements que j'ai déposés -de ne pas oublier les radios associatives et locales ni l'aide aux documentaires. Le système de financement de la création audiovisuelle que tant de pays nous envient est vertueux. Il contribue à faire rayonner l'exception culturelle française ! Continuons à le défendre ensemble. Pour cela, transposons sans perdre de temps les directives SMA et droits d'auteurs,

en augmentation de 8 millions d'euros. J'espère néanmoins que les pouvoirs publics s'investiront davantage pour peser dans les négociations ouvertes avec Google afin d'appliquer la loi dont je suis l'auteur sur les droits voisins en faveur des éditeurs et- je le rappelle, car elles sont un peu oubliées -des agences de presse. D'ailleurs, j'espère que mon amendement, voté par le Sénat, visant à ramener la TVA des productions d'agences de presse de 10 % à 5,5 % ne sera pas annulé par l'Assemblée nationale. Mais à quoi bon une telle aide à la presse si c'est pour, parallèlement, tenter de la mettre sous contrôle avec l'article 24 du projet de loi « sécurité globale » ou l'article 25 de la loi dite loi dite « contre les séparatismes », et même en rendant possible la censure par une circulaire fortement contestée du ministère de l'intérieur ? En s'attaquant à la loi de 1881, au-delà de la presse, c'est la liberté d'expression tous les citoyens dans notre pays que l'on touche. Car comme le déclarait Victor Hugo dès 1848 : « [ ...] Le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. [ ...] Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

Ils ont mis à profit ces moments pour lire les derniers succès de librairie, relire les grands classiques, redécouvrir des films cultes, regarder les dernières séries, télécharger- légalement -les films récents

Les librairies, les disquaires, les bibliothèques, les cinémas, les théâtres, ces lieux où nous avons l'habitude de nous retrouver pour partager des moments si particuliers ont disparu de notre quotidien. Ces adresses, ces commerces, ces salles, nous avons l'obligation de les accompagner financièrement pour qu'ils soient encore en activité après la crise. Pour certains métiers, la crise est bien antérieure à mars 2020,

La consultation de journaux ou d'articles en ligne ou sur des applications s'est évidemment accélérée pendant le confinement, mais cela n'a pas permis de compenser la baisse des ventes papier.

Même si tout n'est pas parfait, Les Français continuent de lire et d'acheter des livres. L'enjeu est de sauvegarder le réseau des détaillants, en d'autres termes les libraires. Leur fermeture fut à juste titre incomprise pendant le second confinement. Le a permis de légèrement limiter l'impact, mais ce sont les géants de la vente en ligne qui ont massivement pris le relai pendant cette période. sont proposées en faveur de ce secteur, c'est une bonne nouvelle, mais une grande vigilance s'impose. Nous devons collectivement bâtir les outils qui permettront de contenir la montée en puissance de certains GAFA, qui sont en train de remettre en cause des modèles qui fonctionnaient plutôt bien

Madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette année 2020 a été très dure pour les médias et les industries culturelles. Les moyens attribués à ces secteurs sont essentiels pour la démocratie, la citoyenneté et l'expression du pluralisme,

La récente création du Centre national de la musique, doté d'importants moyens supplémentaires, va permettre de soutenir fortement le monde de la musique, très impacté par la fermeture des salles de concert. Cependant, madame la ministre, nous vous demandons de rester vigilante sur la répartition de ces aides, afin de ne pas favoriser certains types de musique plus que d'autres. Je pense particulièrement aux musiques actuelles et électroniques, qui peinent à entrer dans les cases, alors qu'elles représentent près de 18 % du chiffre d'affaires de la musique. Il est indispensable de soutenir toutes les musiques sans distinction pour conserver la diversité musicale française. Concernant le programme 180, les efforts budgétaires consentis à la presse et aux médias sont plus que bienvenus. Nous saluons aussi les aides accordées à la presse en ligne. Une refonte de ces aides apparaît toutefois plus que nécessaire,

Parallèlement, les radios locales et associatives ont grand besoin de soutien. La crise sanitaire accentue leurs difficultés alors que leurs recettes étaient déjà en baisse constante.

C'est là que le bât blesse. Comment réussir à prendre le tournant du numérique avec de fortes contraintes de baisse de budget ? Comment atteindre l'objectif de renforcer l'audience chez les jeunes tout en programmant l'arrêt de France 4 ? Comment proposer une offre diversifiée et de proximité France 3 ou France Bleu alors que France Télévisions et Radio France sont contraints à une diminution de 20 % de leurs effectifs d'ici à 2023 ? Nous regrettons également la fermeture des antennes locales de FIP à Bordeaux, Nantes et Strasbourg, alors que l'on connaît leur rôle dans la promotion de la vie culturelle de proximité.

par ailleurs à saluer tous les employés de France Télévisions et de Radio France, mais aussi d'Arte, qui, malgré de fortes contraintes budgétaires, arrivent encore à proposer des programmes de qualité et à conforter leurs audiences. Ils arrivent à faire plus alors qu'on leur donne toujours moins. ce rythme de coupes budgétaires, je ne vois pas comment l'audiovisuel public parviendra à maintenir cette qualité de programmes. Le groupe écologiste dénonce aussi l'arrêt de la diffusion de France Ô. Les habitants des départements et territoires d'outre-mer représentent 3,26 % de la population française. Pourtant, aujourd'hui, ils ne sont plus visibles qu'à 0,4 % sur le service public télévisuel. Le compte n'y est pas ! Le constat est le même pour la représentation des femmes et des minorités. Il est indispensable d'instaurer plus d'obligations légales contre toutes les discriminations et de mener une politique qui va dans ce sens. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera le budget de la mission « Médias, livre et industries culturelles », même si nous craignons qu'il reste insuffisant pour permettre de faire face au contrecoup de la crise sanitaire. En revanche, considérant le manque d'ambition pour l'audiovisuel public, il ne votera pas le budget du compte spécial. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, la crise sanitaire a plongé dans le noir nos cinémas, nos librairies et presque toute notre industrie culturelle. En juillet dernier, les pertes étaient déjà estimées à 22,3 milliards d'euros, un montant que le nouveau confinement va hélas ! aggraver. Au-delà des enjeux économiques évidents que porte la mission, c'est tout un pan de la création culturelle, un marqueur fort de l'ADN de la France, qui est menacé. Certes, nous savons que pour tous ces secteurs, la pandémie ne fait qu'accélérer des difficultés structurelles qui existaient auparavant, des difficultés le plus souvent liées à leur adaptation à la révolution numérique. Néanmoins, les conditions actuelles d'une crise sans précédent doivent vous interroger sur la poursuite des réformes de rationalisation engagées, en particulier au sein de l'audiovisuel public. Celles-ci ne doivent pas prendre un tour brutal, notamment pour les salariés. Avant tout, c'est d'un effort financier exceptionnel qu'ont besoin les entreprises de l'industrie culturelle, qui génèrent des milliers d'emplois. Les mesures transversales, notamment le chômage partiel étendu aux intermittents du spectacle, ont permis d'amortir le choc. Mais cette situation sera-t-elle encore tenable avec les nouvelles jauges proposées aux cinémas et salles de spectacle pour leur réouverture prochaine ? Nous devons reconnaître cependant que les moyens supplémentaires sont au rendez-vous. En effet, s'agissant des seuls crédits de la mission, ils sont en hausse de 8,4 % en autorisations d'engagement et de 3,36 % en crédits de paiement. Par ailleurs, le budget initialement prévu pour 2021 sera renforcé par des sommes représentant 75,3 % de crédits supplémentaires. Tout cela est considérable. Tous les secteurs en bénéficieront, même s'il convient de mettre à part l'audiovisuel public. Nos collègues rapporteurs l'ont souligné : le secteur fait l'objet d'un mouvement contradictoire, avec une baisse de 68,5 millions d'euros des concours financiers à l'audiovisuel public, mais un renfort de la mission « Plan de relance » à hauteur de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 65 millions en crédits de paiement. Cela semble sous-tendre la poursuite de la rationalisation des moyens que vous demandez depuis 2018 aux six sociétés audiovisuelles publiques. Mais, dans ces conditions, il aurait été souhaitable que la réforme de l'audiovisuel ne soit pas remisée. En effet, le choix de mini-contrats d'objectifs et de moyens pour 2020-2022 ne suffira pas à répondre aux enjeux du secteur, qui sont nombreux. Je citerai en particulier le caractère injuste de la contribution à l'audiovisuel public, l'absence de gouvernance commune des entreprises, qui écarte de fait les possibilités de mutualisation, ou encore la concurrence féroce des plateformes américaines au sein de notre paysage audiovisuel. À tous ces défis, il faut apporter des réponses dans ce même temps que l'urgence sanitaire. Je profite de cette discussion générale pour vous interpeller, madame la ministre, sur le sort des télévisions locales, qui rencontrent également des difficultés financières lourdes. J'avais déposé en première partie un amendement d'appel sur ce sujet. Vous savez combien ces médias valorisent les territoires en diffusant des informations de proximité qui intéressent vivement nos concitoyens. Nos collectivités locales les soutiennent, mais cela ne suffira pas à compenser la perte de leurs recettes publicitaires due à la crise sanitaire. Il vous faut agir vite. Concernant la vie de nos territoires, je m'inquiète également de l'avenir de nos librairies et de nos libraires, qui sont des acteurs culturels importants de nos centres-villes, mais aussi de nos centres-bourgs. Beaucoup de ces commerces ont été fragilisés par des mois cumulés de fermeture.

Mais la concurrence redoublée de la vente en ligne par les grandes plateformes depuis le confinement nécessite une réflexion plus large sur la façon de les aider à s'approprier la révolution numérique plutôt que de la subir. S'agissant des auteurs, sur lesquels se répercutent à la fois la fermeture des librairies et l'annulation des événements littéraires, je me réjouis d'un premier soutien de 5 millions d'euros par le biais du Centre national du livre Mes chers collègues, compte tenu de l'effort budgétaire conséquent que porte le projet de loi de finances en direction des médias, du livre et des industries culturelles, le RDSE approuvera la mission, tout en appelant à la poursuite des réflexions et des réformes nécessaires à la préservation de tous les outils qui sont au coeur de la diversité culturelle française. Je veux remercier Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, une enquête de septembre du ministère de la culture estime que les pertes engendrées par la pandémie de coronavirus pourraient, dans le secteur culturel, se chiffrer à près de 23 milliards d'euros. Depuis lors, notre pays a fait face à un second confinement, au moment même où de timides reprises voyaient le jour. Les annonces de jeudi dernier constituent une bouffée d'air frais, même si plusieurs éléments doivent encore être précisés. Le revenu minimal de 900 euros par mois entre novembre et février est-il calibré pour les intermittents, au vu de la conditionnalité imposée ? Dans le même registre, l'année blanche instaurée ce printemps va-t-elle être prolongée pour prendre en compte les nombreuses annulations des prestations prévues au second semestre ? Le soutien de l'État à ces filières en crise n'en demeure pas moins réel, et nécessaire pour les faire survivre. Est-il pour autant suffisant ? Plusieurs inquiétudes demeurent. Premièrement, et comme je l'ai indiqué, il semble que le soutien financier ait été calibré pour le premier confinement. De plus, si des crédits massifs sont inscrits dans la mission et le plan de relance, la baisse des recettes fiscales irriguant les structures nous inquiète tout particulièrement. Deuxièmement, plusieurs actions nous laissent circonspects. Tout d'abord, s'agissant des industries culturelles et du livre, le maintien de la subvention au CNL nous interroge. Le secteur a connu un rebond salutaire durant l'été, mais l'automne devrait être aussi cataclysmique que ce printemps. Et encore, ce regain estival a surtout concerné les auteurs et autrices déjà installés, les éditeurs ayant repoussé les sorties de premiers romans pour éviter qu'ils ne soient étouffés par les plus attendus. Ensuite, je ne ferai qu'évoquer la question du cinéma, déjà abordée dans ma précédente Je m'interroge sur le manque de soutien apporté aux vidéastes hors cinéma. Ces nouveaux créateurs, encore peu considérés par l'État, subissent la crise, alors que leur phase de professionnalisation n'est pas tout à fait aboutie. Cela est d'autant plus problématique qu'ils occupent une place importante dans la lutte pour la démocratisation de l'accès à la culture et la lutte contre les fausses informations, au vu de leurs audiences. Troisièmement, deux points noirs subsistent, les aides à la presse et l'audiovisuel public. Pour le premier secteur, l'augmentation des aides à la presse est salutaire, mais largement insuffisante, pour deux raisons. Tout d'abord, elle ne compense pas les baisses drastiques opérées cette année. Ensuite, le secteur a particulièrement souffert de la crise sanitaire, couplée à sa crise structurelle. Nous ne sommes pas à l'abri de voir des titres disparaître, alors même qu'on voit l'importance de leur rôle dans le bon fonctionnement de la démocratie. En dehors même de cette question du montant des aides, nous devrons réinterroger notre modèle d'aide à la presse, qui, aujourd'hui, ne favorise pas la création d'un pluralisme, tant les médias sont rongés par la concentration. À ce titre, le plan de filière que vous promouvez risque de s'assimiler une nouvelle fois à un afflux d'argent public auprès d'agents économiques opérant des coupes drastiques parmi leurs effectifs. Pour le second secteur, vous nous demandez presque de nous réjouir que la baisse des crédits soit non pas de 80 millions d'euros, mais uniquement de 70 millions d'euros. Pourtant, nous avons encore une fois besoin d'un véritable service public audiovisuel ambitieux, et le maintien pour un an de France 4 n'est qu'un répit. De la même manière, la compensation à hauteur de 70 millions d'euros de la perte des revenus publicitaires

Madame la ministre, on ne peut pas en même temps vouloir l'exigence de l'audiovisuel public, saluer son rôle lors de la crise sanitaire et lui couper les vivres. Qu'on estime qu'il faille une réforme en profondeur de son financement, c'est une chose. Mais, en l'état actuel des choses, rien n'est proposé pour compenser les pertes dues aux décisions gouvernementales. Les pistes proposées par la réforme avortée de votre prédécesseur étaient pour partie insatisfaisantes, notamment en ce qui concerne la publicité, mais avaient le mérite d'exister. Quel plan a le Gouvernement aujourd'hui pour un réinvestissement du service public audiovisuel ? En conclusion, certains pans de ce budget sont satisfaisants et témoignent d'un réel investissement du Gouvernement. On peut citer, comme je l'ai fait tout à l'heure, le cinéma. Malheureusement, d'autres secteurs comme la presse et l'audiovisuel public sont mis au ban.

Mon intervention portera sur l'ensemble du champ de la mission, à l'exception notable des crédits de l'audiovisuel et de la chaîne du cinéma, dont parlera notre collègue Catherine Morin-Desailly. À l'instar de tous les secteurs culturels, la presse a bien sûr énormément souffert de la crise sanitaire. Notre rapporteur, Michel Laugier, dont je salue au passage l'excellence du travail, vient de rappeler les chiffres : la diffusion a diminué de 20 %, les recettes publicitaires de 80 %. C'est un séisme, surtout pour un secteur dont les difficultés sont antérieures à la crise de la covid, et qui doit subir par ailleurs le double choc de l'émergence du numérique et de la faillite de Presstalis. Avec notre commission, nous ne pouvons donc que saluer le maintien de l'effort de soutien au secteur, de même que les avancées positives dans la reconnaissance de la presse en ligne, la création du fonds de lutte contre la précarité dans la profession de journaliste et sur le dossier clef des droits voisins. Depuis le début de la crise, la situation du livre, celle des librairies, est sous le feu des projecteurs. Et pour cause, elles auraient dû, selon nous, rester ouvertes. À notre connaissance, les librairies n'ont jamais été des clusters. Or le présent budget ne traduit pas l'inquiétude exprimée dans l'opinion publique à leur sujet. En effet, le soutien à la filière ne fait pas l'objet d'une augmentation de crédits au sein de la mission. Seul le plan de relance concrétise un soutien financier ponctuel, mais un soutien mesuré : sur les 370 millions d'euros consacrés au secteur culturel, seuls 30 millions d'euros doivent aller au livre. C'est peu. Heureusement, les librairies ont bénéficié après le premier confinement d'un effet rebond. Nous espérons que le phénomène se reproduira pour les fêtes de fin d'année. De plus, même si le ne remplacera jamais une activité normale, les commandes en ligne ont pu permettre aux librairies de sauvegarder un minimum d'activité, entre 20 % et 30 %. La situation de la Bibliothèque nationale de France est à surveiller. En effet, bien que ses crédits soient en hausse continue ces dernières années, les grands et ambitieux projets dans lesquels elle s'est lancée, ainsi que la crise sanitaire, pourraient à terme fragiliser son équilibre financier et entamer sérieusement ses marges de manoeuvre. Le recours au mécénat, que je salue ici, ne doit cependant pas se substituer graduellement au soutien de l'État. La situation des salles de cinéma est tout autre. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à abonder de 70 millions d'euros l'action Culture dans le plan de relance. Nous regrettons fortement qu'il n'ait pas été adopté. En effet, depuis le début de la crise, le manque à gagner pour les salles de cinéma avoisinerait déjà le milliard d'euros. Une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros a été débloquée en LFR 3 pour le dernier trimestre 2020, mais le plan de relance est très sous-dimensionné pour prendre le relais de cette aide. Seuls 37 millions d'euros sont prévus pour les salles en 2021. Le risque est grand de les voir mourir. Même lorsqu'elles pourront rouvrir, les salles vont souffrir d'un effet psychose persistant. La jauge à 50 %, avec une place sur deux, et le port du masque tout au long du film pourrait aussi faire s'envoler l'effet « détente » d'une séance de cinéma. Vous le savez, mes chers collègues, les salles de cinéma sont l'un des maillons essentiels de l'écosystème de la création cinématographie dans notre pays. Si les salles disparaissent, c'est toute la filière qui sera menacée. Il y aura toujours des producteurs pour faire des films, mais s'il n'y a plus personne pour les diffuser, c'est l'industrie entière qui perd sa base. Sans oublier non plus toute l'importance des cinémas dans l'animation culturelle et artistique de nos territoires. J'en terminerai par le secteur de la musique, dont la situation est, elle aussi, très préoccupante hélas ! Heureusement, le soutien financier qui lui est accordé n'est pas négligeable. Le Centre national de la musique a reçu 50 millions d'euros en LFR 3 et va recevoir 200 millions d'euros, soit treize fois sa dotation, pour mettre en place le soutien à la filière musicale dans son ensemble- spectacles, concerts et musique enregistrée. Ce soutien compensera notamment les pertes de billetterie. Plusieurs points de vigilance sont toutefois Une institution si jeune sera-t-elle en mesure d'accomplir une telle mission ? Par ailleurs, malgré l'effort, ce soutien sera sans doute lui aussi insuffisant. Pour le compléter, nous proposerons dans les articles non rattachés un amendement exonérant de cotisation foncière des entreprises (CFE) les TPE de musique enregistrée et d'édition musicale, ce qui devrait profiter à toute la chaîne de production musicale. Enfin, le présent PLF consacre la montée en charge des crédits propres au CNM, qui doit prendre pleinement ses fonctions en 2021. Sa subvention atteint presque 16 millions d'euros. C'est conforme aux engagements gouvernementaux, mais le financement pérenne du CNM n'est toujours pas assuré. C'est un dernier point de vigilance.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la pandémie marque un véritable tournant pour le monde de la culture. Pour autant, cette pandémie n'est pas à l'origine- il s'agit bien d'un choix du Gouvernement -du report de la réforme tant attendue de l'audiovisuel public, alors même que l'année 2020 devait être la grande année de la réforme de sa gouvernance et de son financement. Pour les deux prochaines années, les Français continueront de s'acquitter d'une CAP qui n'est plus représentative des usages du numérique. Les multiples initiatives des opérateurs sont pourtant la preuve de leur volontarisme, au service d'un audiovisuel public fort, qui se réinvente pour réaffirmer sa spécificité. filière mérite donc d'être soutenue par un nouveau cadre législatif et réglementaire, adapté à l'essor du numérique et à la véritable explosion d'offres venues bouleverser le marché mondial. En ce sens, nous ne pouvons que nous réjouir de la transposition de la directive SMA, qui crée les conditions d'un nouveau partenariat équilibré avec les services de vidéo à la demande.

La prise en compte de la spécificité des plateformes, la nature de leurs catalogues, leur place dans la chronologie des médias et la répartition des visionnages entre audiovisuel et cinéma laissent entrevoir une modernisation utile et positive de la politique audiovisuelle, dont nous pouvons tous nous réjouir. Pour 2021, les moyens alloués à l'audiovisuel public suivent, comme l'an dernier, une trajectoire financière déclinante, résultant de l'objectif de réduction de 190 millions d'euros sur la période 2018-2022. En dépit des 70 millions d'euros prévus par le plan de relance, l'effort budgétaire demandé aux opérateurs est trop important dans le contexte difficile de crise sanitaire que nous connaissons, et au vu des pertes importantes de recettes publicitaires.

En ce qui concerne France Médias Monde, en tant que membre du conseil d'administration, je peux attester de son rôle à l'international et des efforts fournis par la direction afin d'améliorer la situation financière de l'entreprise, au travers du plan de départs volontaires voté en 2019. Les contrats d'objectifs et de moyens, bien que ne compensant pas l'absence de gouvernance commune, permettront aux six opérateurs de défendre cinq objectifs communs : la mise en avant de la singularité de l'offre publique, la mutualisation des achats, la concentration des moyens vers l'offre au public et la variété des programmes, la stabilité financière et l'exemplarité sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, de réduction de l'empreinte carbone, d'insertion dans l'emploi et de défense de la laïcité. Sur ce dernier point, cette année 2020 est particulièrement difficile pour notre audiovisuel extérieur. France Médias Monde et TV5 Monde ressentent en effet pleinement les tensions internationales réveillées par la réaffirmation de l'attachement indiscutable de la France à la défense de la liberté d'expression. En ce qui concerne les industries culturelles, le cinéma a été impacté à tous les niveaux des chaînes de production et de distribution et a subi un véritable coup d'arrêt. En temps de crise, ce sont les plus petites structures qui sont le plus souvent touchées, en l'occurrence le cinéma indépendant. La mission « Plan de relance », qui prévoit 165 millions d'euros en faveur du cinéma, devrait, comme le souligne le rapport de la commission des finances, permettre de compenser un effondrement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en 2020. Dans le même temps, elle permettra de financer les crédits dédiés aux dispositifs mis en place en faveur d'un rebond de l'industrie cinématographique. Dans ce contexte difficile, sans aucune visibilité, il convient de saluer l'action du CNC en faveur d'un rebond rapide du secteur, selon trois axes clefs : rattraper le retard de production, encourager la sortie des films en période de reprise et assurer la viabilité des salles de cinéma à court et à long terme. Cette année marque également l'entrée en fonction du Centre national de la musique. En plus des missions qui lui avaient été confiées, le CNM s'est retrouvé en première ligne pour sauver un secteur dont le pronostic vital était engagé. Je salue le dévouement dont ont fait preuve les équipes, ainsi que le maintien des crédits qui lui avaient été alloués. Je m'associe à la proposition du rapporteur spécial de voir réaliser un bilan d'activité du CNM, dans un rapport dédié, au terme de cette première année d'existence. Toutefois, le secteur de la musique, dans son ensemble, n'a pas été assez pris en compte et nous nous en inquiétons. Ce sera un point de vigilance particulier. Enfin, je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble de ces acteurs qui, en période de crise, n'ont cessé d'oeuvrer pour maintenir leur secteur à flot, au service de l'exception culturelle française. Nous ne pouvons que nous incliner devant leur résilience. Hormis les réserves exprimées, mes chers collègues, notre groupe s'en remettra à l'avis de nos rapporteurs et votera pour l'adoption des crédits de la mission et ceux du compte spécial dédié à l'audiovisuel public. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la présidente,

Madame la présidente, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, oui, 2020 aurait dû être enfin l'année de la réforme audiovisuelle promise par le Président de la République ! Après des débuts laborieux, Franck Riester l'avait remise sur les rails ; voilà que la crise sanitaire est le prétexte à tout abandonner

face à une concurrence extraeuropéenne exacerbée, nous pouvons nous interroger, d'un point de vue stratégique, sur la baisse continue des moyens affectés à notre audiovisuel public depuis 2018. Cette année, la trajectoire est stable et, point de satisfaction, est assortie d'une dotation exceptionnelle pour répondre à la crise sanitaire, bien que la réponse doive être nuancée en fonction des opérateurs- j'y reviendrai. Les chiffres et les coups de communication sont louables, mais nous avons aussi besoin d'une vision d'avenir. Quelle stratégie, quelle réponse structurelle adopter pour donner à nos médias les moyens d'une alternative à la standardisation d'une offre de plus en plus globale et anglo-saxonne ? L'ensemble du secteur de la création audiovisuelle et cinématographique est concerné, les chaînes, publiques comme privées, étant soumises à des obligations en matière d'investissement. Nous veillerons aux équilibres entre les acteurs de la chaîne médiatique dans le futur décret de transposition des directives. La manière dont nos entreprises audiovisuelles ont fait preuve d'adaptabilité et de résilience face à la crise ne doit pas cacher leur fragilité structurelle et budgétaire. Voyez la chute des recettes publicitaires Plus que jamais, les modèles sont à clarifier et la réforme de la CAP à mener, ne serait-ce aussi que parce qu'elle est profondément injuste. Sur ce point, nous insisterons toujours sur la nécessité d'une dotation publique et non d'État, seule garante de la véritable indépendance. Objectifs et missions doivent être reprécisés. Personne n'a compris la suppression de France Ô et de France 4, présentée strictement sous l'angle budgétaire et non sous celui des besoins des publics. Quel sera l'avenir de la chaîne jeunesse temporairement réhabilitée ? La stratégie est-elle de désarmer l'audiovisuel public face à Disney et YouTube ? En l'état du réseau, tous les Français ne reçoivent pas Okoo. France 4, désormais dépourvue de publicité grâce au Sénat, pour laquelle mon ancien collègue Jean-Pierre Leleux et moi-même avions déposé un moratoire, a démontré à quel point elle était un outil indispensable à l'éducation, à la culture et à la citoyenneté. Interrogé devant notre commission, Jean-Michel Blanquer lui-même est convenu de la nécessité de son maintien.

Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'offensive d'Al Jazeera à la suite à l'assassinat de Samuel Paty. Alors que France Médias Monde aurait dû être renforcée- nous ne cessons de le dire ici, année après année -, voilà que l'entreprise est contrainte à des arbitrages douloureux entre nouveaux projets nécessaires et préservation des zones de diffusion. La chaîne franco-allemande Arte, qui est de plus en plus européenne et innovante, enregistre toujours une baisse de la ressource publique.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, suite de l'année que nous venons de vivre et de l'épidémie de covid-19 qui a bouleversé tant de secteurs, je tenais à saluer la formidable capacité d'adaptation et de résilience de notre audiovisuel extérieur, tant France Médias Monde que TV5 Monde, dont les personnels ont, par leur dévouement et leur professionnalisme, fait honneur à l'audiovisuel public.

mais aussi en contribuant au service public d'éducation- je pense à Radio France internationale (RFI), qui a proposé « L'école à la radio » -notre audiovisuel extérieur a montré toute son implication et le rôle stratégique qu'il pouvait jouer. Ce rôle a été justement plébiscité par le public, puisque toutes les chaînes ont vu leurs audiences sensiblement augmenter. Compte tenu de cet apport, nous ne pouvons que regretter que France Médias Monde et TV5 Monde ne reçoivent que 500 000 euros chacune sur les 70 millions d'euros du plan de relance consacré à l'audiovisuel public. Nous ne pouvons également que regretter que la dotation attribuée à France Médias Monde dans le PLF 2021 soit en recul de 0,5 million d'euros par rapport à l'année dernière, et que celle de TV5 Monde soit stable- seulement stable alors même que la France occupe pour 2020-2021 la présidence tournante de la chaîne. Malgré cette trajectoire financière peu ambitieuse, nous devons nous féliciter de la poursuite par France Médias Monde de sa dynamique de progression mondiale et de développement de projets ambitieux, comme la diffusion de France 24 en espagnol, qui touche désormais 6,8 millions de foyers. La coopération audiovisuelle franco-allemande doit également être saluée à sa juste mesure, tant le partenariat entre France Médias Monde et la est porteur d'espoir pour raviver l'idéal européen et lutter contre les populismes et la désinformation. la ministre, je souhaitais partager mon inquiétude sur la diminution des ressources commerciales- publicitaires notamment -qui touche France Médias Monde et TV5 Monde, à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19. Compte tenu du fait que ces ressources devraient continuer à diminuer en 2021, il sera nécessaire d'être vigilant sur ce point et de soutenir notre audiovisuel extérieur, pour qu'il continue dans la mission stratégique qui est la sienne.

Madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour le secteur des médias, presse, livre et industries culturelles, l'année 2020 aura été dévastatrice. Les orateurs précédents l'ont répété. Au mois de juillet dernier, avant même l'annonce du reconfinement le 28 octobre, le ministère de la culture évaluait les pertes de chiffre d'affaires du secteur des médias et des industries culturelles à 22,3 milliards d'euros. Les plans d'urgence et les fonds de secours sectoriels se sont succédé jusqu'au projet de loi de finances. Cette cascade de financements, les uns urgents, les autres relevant de la classique discussion budgétaire, rendent l'exercice d'analyse plus complexe, mais néanmoins nécessaire. Concernant la presse, si je salue le soutien continu apporté aux différents acteurs de la filière, dans le prolongement du sauvetage de Presstalis, je ne comprends toujours pas pourquoi la presse professionnelle, celle de la connaissance et du savoir, est systématiquement écartée des aides, alors que la presse d'information politique et générale Aussi, je souhaiterais que mon amendement instituant un crédit d'impôt pour un premier abonnement à l'un de ces titres puisse être conservé dans la loi de finances. Concernant la musique et le spectacle vivant musical, le soutien qui lui est apporté le Centre national de la musique est significatif, en complément du fonds de secours destiné aux PME et TPE du secteur. Néanmoins, un vrai problème demeure, celui de la diminution des aides à la création allouées par les organismes de gestion collective, dans un contexte marqué par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2020, qui divise par deux les « irrépartissables Cela représente une perte de 25 millions d'euros par an pour la diffusion du spectacle vivant ou la formation des artistes. Le cinéma est également un secteur de la culture très sinistré. Pour le soutenir, j'ai déposé plusieurs amendements instituant des crédits d'impôt ou élargissant l'assiette de ceux qui existent.

Enfin, j'insisterai sur le secteur du livre, qui me tient particulièrement à coeur. La fermeture des librairies était- je le dis tout net -une erreur majeure. La forte mobilisation des professionnels et des élus a d'ailleurs démontré l'attachement à ce service de proximité essentiel, vecteur de lien social et lieu de diffusion de la culture, du savoir et de la connaissance. J'ajoute que l'on ne pouvait décemment croire que le « cliquer et collecter » était à lui seul de nature à sauver les librairies, de même que l'allégement des tarifs postaux, qui devront impérativement être pérennisés. Il faut néanmoins saluer les efforts d'accompagnement mis en place en leur faveur dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 : par l'intermédiaire du Centre national du livre, 25 millions d'euros ont été alloués aux librairies pour soutenir leur trésorerie et 6 millions d'euros pour la modernisation de leur outil numérique. millions d'euros ont par ailleurs été fléchés vers les maisons d'édition. Les auteurs et les artistes ont, quant à eux, pu accéder au fonds de solidarité, mais ils n'y étaient pas tous éligibles lors de sa mise en place, à défaut de disposer d'un numéro Siret. Je me réjouis que l'amendement de notre collègue Sylvie Robert et le mien, visant à défiscaliser et désocialiser les aides qui leur ont été versées par les fonds d'urgence sectoriels, aient été satisfaits. Concernant le livre et la lecture, le budget 2021 progresse, mais cette augmentation correspond en grande partie au soutien consenti à la Bibliothèque nationale de France pour la réhabilitation du site Richelieu et le financement adéquat de ses missions. comme pour les autres industries culturelles, vous avez également décidé, madame la ministre, de présenter un plan « filière livre », soutenu par les crédits du plan de relance et orchestré par le CNL, à hauteur de 29,5 millions d'euros en crédits de paiement et 53 millions d'euros en autorisations d'engagement. Que l'État accentue son soutien en faveur des collectivités territoriales, en modernisant leurs bibliothèques et en renforçant leur budget d'achat de livres imprimés auprès des librairies de proximité, est une excellente nouvelle. C'est un moyen de développer la pratique de la lecture chez nos concitoyens, notamment les plus jeunes, qui bénéficieront de la distribution de chèques « Lire de la distribution de chèques « Lire ». La poursuite de l'aide à la modernisation de l'outil numérique des librairies, qui sera doublée, après l'enveloppe de 6 millions d'euros déjà ouverte dans la troisième loi de finances rectificative, Toutes ces mesures indispensables permettront-elles cependant à l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, imprimeurs et distributeurs, de surmonter les conséquences des deux confinements et de prendre de nouveau des risques pour promouvoir la diversité culturelle française ? Tous les grands événements autour du livre et de la lecture, notamment les salons et manifestations, attendus chaque année par les lecteurs, ont dû être annulés. Quelle tristesse de voir cette semaine les grands prix littéraires proclamés par visioconférence, même si je félicite chaleureusement les lauréats Je veux toutefois être optimiste : continuons à défendre ces enjeux essentiels pour notre pays que sont la vitalité culturelle, la diversité de la création, le rayonnement des idées et la diffusion des oeuvres de l'esprit. Je sais pouvoir compter sur votre engagement personnel, madame la ministre. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera les crédits de cette mission. La parole

mes chers collègues, depuis le mois de mars, nous vivons dans l'incertitude la plus totale. La peur du coronavirus s'est installée chez chacun d'entre nous. Nous avons alors ressenti un immense besoin d'information. Le décryptage de l'épidémie par les médias et par leurs consultants spécialisés a été très suivi par les Français. L'accès à des données fiables sur la situation sanitaire, économique et sociale de notre pays était souhaité et recherché dans tous les médias. Depuis que nous sommes confinés, nous avons aussi pris conscience du caractère fondamental des relations humaines et de la culture, vecteur de découvertes et d'évasion, échappatoire en période de pandémie. Les secteurs des médias, du livre et des industries culturelles se sont imposés à nous comme essentiels. Malheureusement, ils font surtout partie des secteurs les plus fragilisés par la crise. En effet, depuis le mois de mars, les auteurs n'ont plus la possibilité d'intervenir ni de défendre leurs titres. Les librairies et les médiathèques ont fermé, puis testé le. Le transport Le transport des livres a été fortement ralenti. Les éditeurs ont perdu la plus grande partie de leurs interlocuteurs et les sorties ont dû être reportées. Les manifestations ont été annulées, ou reportées, et dans quelques cas proposées en version numérique. Il est possible que cette période exceptionnelle fasse naître aussi des chefs-d'oeuvre d'artistes inspirés par la crise. Toutefois, comment ces ouvrages seront-ils diffusés dans notre pays sans des maisons d'édition et des librairies en bonne santé économique ? Le confinement a mis un coup d'arrêt au monde des livres, et la crise a montré toute la difficulté, notamment pour les librairies indépendantes, de faire face de faire face au numérique et de s'adapter aux nouveaux modes de consommation des Français. Ces lieux, si chers à nos centres-villes, doivent être soutenus, afin qu'ils ne ferment pas définitivement, mais aussi afin qu'ils s'engagent, enfin, dans le numérique. L'enjeu est de taille et le défi urgent à relever, car les jeunes générations s'éloignent des commerces physiques au profit des plateformes de commerce en ligne. Elles s'éloignent également du format papier pour préférer le format numérique les ventes de liseuses électroniques ont connu une belle embellie, dès le premier confinement, avec jusqu'à 130 % de ventes supplémentaires. Le déconfinement et l'été n'ont pas freiné la tendance. Si les grands acteurs du livre s'en accommodent, les librairies indépendantes ne vont pas avoir d'autre choix que de s'adapter à ce nouveau marché et de devenir, elles aussi, un acteur dans le développement de ces nouvelles manières de lire. de lire. Qu'en sera-t-il pour tous les imprimeurs, distributeurs, diffuseurs, qui voient leur modèle économique mis en jeu ? Leurs craintes pour l'avenir sont grandes et légitimes. En 2021, le programme 334, « Livre et industries culturelles », atteindra 317 millions d'euros. Le secteur bénéficiera de 10,8 millions d'euros de moyens supplémentaires pour répondre à ces enjeux culturels incontournables. Dans cette démarche, l'État peut et doit s'appuyer sur les agences régionales du livre et de la lecture pour soutenir tous les acteurs du secteur. Dans les Hauts-de-France, par exemple, l'agence régionale du livre et de la lecture met en réseau les professionnels et fait un travail remarquable pour les accompagner et développer l'accès du livre et de la lecture pour tous.

mes chers collègues, le décès de l'ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing a été annoncé ce soir. Il reviendra au Président Larcher d'organiser l'hommage que le Sénat lui rendra.

monsieur le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, monsieur le rapporteur spécial, madame, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, tout d'abord, je veux m'associer à l'émotion qui a envahi votre Haute Assemblée à l'annonce du décès du Président Valéry Giscard d'Estaing, et saluer avec vous sa mémoire. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel et c'est la fin de la tutelle de l'Office de

en progression de 3,2 %, ce qui va donc cranter le prochain budget. La mission comportera 19 millions d'euros de moyens nouveaux, dont bénéficieront l'ensemble des filières, en particulier la presse, le livre, l'audiovisuel et le cinéma. L'action menée par le ministère de la culture pour accompagner les industries culturelles s'appuiera également sur les financements exceptionnels inscrits dans le cadre du plan de relance, qui s'élèvent à 428 millions d'euros sur deux ans, et dont la majeure partie, à hauteur de 347 millions d'euros, sera mobilisée dès 2021. Je remercie le rapporteur spécial Roger Karoutchi d'avoir parfaitement détaillé ce budget. Au total, l'an prochain, c'est donc plus de 1 milliard d'euros qui seront consacrés aux médias et aux industries culturelles. À ces moyens s'ajouteront 400 millions d'euros sur cinq ans, dans le cadre du quatrième programme d'investissements d'avenir (PIA 4). Ces fonds seront consacrés à la mise en oeuvre d'une ambitieuse stratégie d'avenir pour nos industries culturelles et créatives, qui vise à répondre à notre objectif de réconciliation entre les pratiques culturelles et patrimoniales, ces pratiques étant considérées comme traditionnelles, et les pratiques numériques. Cette mobilisation budgétaire exceptionnelle va nous permettre de soutenir les filières culturelles qui ont été durement touchées par l'application des mesures sanitaires du printemps dernier, et dont certaines pâtissent encore- vous l'avez tous souligné. Je pense en particulier au cinéma, qui, depuis le début de la crise, bénéficie d'un accompagnement spécifique constamment adapté à l'évolution de la situation sanitaire. Au-delà des mesures d'urgence dont ont bénéficié les acteurs de la filière au printemps dernier, nous avons favorisé la reprise d'activité en mettant en place un fonds d'assurance et de garantie financé par l'État à hauteur de 50 millions d'euros, pour que les tournages puissent de nouveau avoir lieu. Depuis septembre, le secteur a bénéficié de 80 millions d'euros d'aides nouvelles destinées en particulier aux distributeurs, aux salles de cinéma, dont la fréquentation a été limitée par l'application des mesures de distanciation physique, puis de couvre-feu. Jérémy Bacchi, vous avez appelé mon attention sur les cinémas en régie directe, qui représentent 400 établissements sur le parc de 6 000 salles. Ce sont des maillons essentiels de la vie culturelle locale, des cinémas dont le modèle économique dépend directement des collectivités territoriales, et qui ne supportent donc pas de risques d'exploitation directs. En raison de cette différence, et par application du principe d'égalité, évidemment, le fonds de compensation cinématographique, créé par l'État et porté par le CNC, n'intègre pas les 400 régies directes. Toutefois, celles-ci bénéficient évidemment de l'intégralité des autres mesures de relance : mesures transversales, mesures spécifiques de renforcement du soutien prévues pour les exploitants de salles de cinéma, soit 30 millions d'euros pour l'ensemble du parc. De plus, j'ai demandé que, sur un certain nombre de sujets spécifiques, si vraiment des salles étaient en très grande difficulté, le CNC puisse, à titre exceptionnel, intervenir. Je voulais donc vous rassurer. Nous continuons à soutenir le cinéma face aux conséquences du confinement et nous serons au rendez-vous pour accompagner la mise en oeuvre du protocole sanitaire et des nouvelles modalités de couvre-feu à partir du 15 décembre. Enfin, pour permettre une reprise durable et pérenne de la filière, le volet culturel du plan de relance comporte une enveloppe de 165 millions d'euros, dont bénéficieront l'ensemble des acteurs Cette aide exceptionnelle s'ajoutera aux ressources habituelles du CNC, qui demeureront, en 2021, relativement stables, jouant ainsi un important rôle contracyclique. Les moyens que nous mobiliserons en 2021 pour les médias et les industries culturelles visent non seulement à répondre aux difficultés immédiates, mais aussi à préparer la reprise. Ils doivent aussi nous permettre de mener un important effort de consolidation et de modernisation des filières culturelles confrontées à des difficultés structurelles qui se sont trouvées exacerbées par la crise sanitaire. En 2021, l'ensemble des programmes de la mission « Médias, livre et industries culturelles » contribueront à ces objectifs, à commencer par le programme « Presse et médias », qui verra son budget progresser de 2,9 %, soit 8 millions d'euros. Cet effort a été salué par Michel Laugier, mais également par Pierre-Antoine Levi. Ces moyens nouveaux et pérennes s'intégreront dans le cadre du plan de filière pour la presse, présenté par le Président de la République le 27 août dernier, et doté de 483 millions d'euros sur la période 2020-2022. Le financement de ce plan de modernisation massif repose en majeure partie sur la LFR 3 de 2020 et le plan de relance, qui apporteront des moyens afin de remédier sur le long terme à une situation de fragilité qui s'aggravait depuis des années. Ainsi, le fonds stratégique pour le développement de la presse sera renforcé, tout comme l'aide à la modernisation des diffuseurs de presse. Des moyens nouveaux seront mobilisés dans le cadre d'un fonds de transformation des imprimeries de la presse régionale, d'un fonds pour la transition écologique et d'un fonds de lutte contre la précarité, qui assureront une meilleure prise en compte d'impératifs absolument fondamentaux pour l'avenir de la filière. Les mesures nouvelles, inscrites dans le PLF 2021, permettront, quant à elles, la mise en place de nouvelles aides au pluralisme, l'une à destination des services de presse en ligne d'information politique et générale, 4 millions d'euros par an, et une autre à destination de la presse ultramarine, pour 2 millions d'euros par an. Elles contribueront ainsi à conforter l'accès de tous nos concitoyens à une information diverse et de qualité sur tous les territoires. Le programme « Livre et industries culturelles » connaîtra également une hausse de ses moyens l'an prochain de 3,5 %, soit 10,8 millions d'euros. y a des mesures à destination de la filière musicale, en particulier le renforcement des moyens du CNM, et, je rassure Monique de Marco, il ne s'agit pas d'exclure de ces mesures les musiques actuelles, dont la musique électronique. Bien entendu, elles font partie des secteurs aidés dans ce cadre. J'ai déjà beaucoup évoqué, lors de l'examen de la mission « Culture », les nouveaux crédits qui financeront l'achèvement du chantier de restauration du site Richelieu de France. J'ajoute que 30 millions d'euros seront également ouverts en autorisations d'engagement pour que la BNF puisse lancer la construction d'un nouveau centre de stockage pour ses documents, lequel devrait être opérationnel d'ici à 2027.

propos. Madame la sénatrice, je suis attachée à Fip, comme à tous les programmes de Radio France. Dans le cadre de son nouveau projet stratégique, Radio France a fait le choix de recentrer Fip sur son programme national, qui forme le coeur de son identité, de sa force prescriptrice, tout en démultipliant la couverture territoriale du programme. Aujourd'hui, Fip est disponible dans seulement dix villes. Désormais, avec le numérique terrestre, elle sera disponible auprès de 85 % de la population. C'est un vrai choix territorial. J'ajoute que cette évolution se fait avec une grande attention portée au personnel, et a fait l'objet de discussions approfondies avec les organisations syndicales. Un accompagnement individuel est ainsi prévu pour les collaborateurs concernés, ce qui est essentiel.

financé par la LFR 3 de 2020 et le plan de relance, dont l'un des grands objectifs est de soutenir l'activité des librairies et des bibliothèques. Laure Darcos et Julien Bargeton en

Cet audiovisuel public continuera en 2021 à respecter la trajectoire décidée en 2018 dans le cadre d'une ambitieuse stratégie de transformation. Ainsi, le compte de concours financiers pour l'audiovisuel public s'élèvera l'an prochain à 3,72 milliards d'euros. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public dont s'acquitteront nos concitoyens restera stable par rapport à l'an dernier, à 138 euros. Afin de tenir compte de la décision que j'ai prise l'an dernier de prolonger jusqu'à l'été 2021 la diffusion linéaire de la chaîne France 4, l'effort d'économies demandé aux sociétés de l'audiovisuel public, qui devait s'élever à 80 millions d'euros, a été réduit de 10 millions d'euros. Je veux dire à Catherine Morin-Desailly qu'il ne s'agit pas de renoncer au rôle d'éducation de la jeunesse assuré par le service public. Il s'agit de réfléchir à un média jeunesse qui ne saurait se résoudre à être une chaîne du confinement. Il faut bien analyser les besoins de la jeunesse dans ce cadre

Parallèlement, afin de compenser les impacts de la crise sanitaire et de préserver la capacité de l'audiovisuel public à investir dans la création, 70 millions d'euros lui seront accordés dans le cadre du plan de relance. saluée sans entrain, j'en conviens, pour reprendre la formule de Jean-Raymond Hugonet, mais l'essentiel est d'être salué ; l'entrain vient en supplément. Je tiens à souligner que cette enveloppe spécifique ne vaut pas annulation de l'effort financier demandé aux sociétés de l'audiovisuel public, mais elle répond à un besoin ponctuel et impérieux lié au contexte de la crise.

Rappelez-vous, en janvier 2019, la France et l'Allemagne ont affirmé leur volonté, dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle, de soutenir le développement d'une plateforme numérique franco-allemande destinée au public jeune et exposant des contenus audiovisuels et d'information. Des travaux de coordination sont en cours avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les diffuseurs et les administrations, afin d'aboutir à une articulation satisfaisante. Ces travaux continuent et ils sont approfondis, mais ils sont retardés par par des dissensions persistantes du côté allemand, liées au partage des compétences dans le champ audiovisuel entre les niveaux fédéral et fédéré.

cafouillage, si l'on peut dire, qu'il convient de régler avant d'avancer, mais notre volonté est toujours extrêmement forte pour faire en sorte que ces dispositions issues du traité d'Aix-la-Chapelle voient le jour. J'y veille. Au-delà du financement pour l'an prochain, une vaste réflexion doit avoir lieu, comme vous le savez, au sujet des ressources de l'audiovisuel public, compte tenu de la suppression totale, à l'horizon 2023, de la taxe d'habitation, à laquelle est adossée la contribution à l'audiovisuel public. Ce travail a déjà débuté, en lien étroit avec le ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt. Je souhaite que nous puissions l'approfondir avec l'ensemble des parlementaires, que je sais très attentifs à ce sujet d'importance tant pour l'audiovisuel public que pour l'équilibre du secteur. L'année 2021 verra également l'aboutissement d'une évolution majeure de notre système de financement de la création audiovisuelle et cinématographique, qui permettra aux acteurs français de ces filières d'accéder à de nouvelles ressources.

! » Vous avez aussi été nombreux à insister sur l'importance de la transposition de ces directives européennes. J'y veille également, selon le calendrier prévu. Vous avez témoigné de votre volonté unanime d'intégrer les plateformes numériques ciblant le public français à notre système de contribution à la création. Céline Boulay-Espéronnier s'est expliquée sur ce sujet. Cette véritable révolution dans le processus de transposition est en cours et sera effective prochainement grâce à l'ordonnance et au décret SMAD. Elle permettra de refonder et restructurer notre modèle en l'adaptant aux nouveaux équilibres entre les acteurs des médias et ceux du numérique. Je souhaite, en effet, que la mise en oeuvre de la directive ouvre la voie à rééquilibrage d'ensemble de notre système de financement de la création, qui passera également par une révision des obligations des chaînes historiques. Des concertations vont d'ailleurs s'engager avec les acteurs concernés.

Pour terminer, je veux donc évoquer, en réponse à ces intervenants, la stratégie d'avenir pour les industries culturelles et créatives, dont j'ai dit quelques mots au début de mon intervention. Financée à hauteur de 400 millions d'euros sur cinq ans, dans le cadre du quatrième programme d'investissements d'avenir, elle sera également soutenue en 2021 grâce aux 19 millions d'euros de crédits inscrits dans le plan de relance. En étant intégrée à ce programme, la culture se trouve pleinement reconnue comme un secteur stratégique, au même titre que l'hydrogène ou les intelligences artificielles. Cette stratégie d'avenir repose sur une démarche inédite, qui rassemblera l'ensemble des filières culturelles, y compris le patrimoine, les arts visuels, le spectacle vivant, autour d'objectifs communs. Les moyens que nous déploierons visent à accompagner les acteurs culturels afin d'accélérer la transition numérique de l'ensemble du secteur et donc de préparer l'avenir. Il s'agira notamment de développer des projets culturels innovants, comme la diffusion de captations de spectacle et le déploiement de nouveaux outils de valorisation du patrimoine, qui offriront de nouveaux moyens de toucher tous les publics. Il s'agira enfin de renforcer la place des acteurs culturels français dans le contexte de forte concurrence internationale, en favorisant le recours à des technologies innovantes. Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont les moyens grâce auxquels le budget de la mission « Médias, livre et industries culturelles », soumis à votre examen, nous permettra de mener l'an prochain une action ambitieuse pour consolider nos filières culturelles, prendre un temps d'avance sur les évolutions à venir et engager une étape décisive de la modernisation de notre politique d'accès à la culture au service de tous les publics. Il est, comme le budget de la mission « Culture », un budget de responsabilité bâti en complémentarité avec le plan de relance, qui apporte des moyens à la hauteur des nombreux défis structurels qui s'imposent au monde de la culture. Je veux remercier les rapporteurs, ainsi que tous les intervenants,

à statut associatif le plus souvent, ont poursuivi et renforcé leurs programmes au bénéfice de leurs auditrices et des leurs auditeurs, des services de l'État, dans des conditions budgétaires dramatiques, aucun geste n'a été fait en leur direction. Pourtant, ils ont été unanimement salués, y compris par le Conseil supérieur Ce travail de terrain lors du premier confinement a permis de maintenir le lien social dans les quartiers, les campagnes, auprès de travailleurs indépendants et des petites entreprises durement impactés. locale (FSER), d'un montant de 1 million d'euros, est prévue pour 2021, mais, comme vous le savez, elle est spécifiquement destinée à compenser l'augmentation du nombre de services autorisés, notamment en radio en radio numérique terrestre, ou DAB. Cette augmentation limitée, qui équivaut à 1 500 euros par radio, ne prend pas en compte l'impact dramatique de la crise sanitaire. Je veux donc plaider dans cet hémicycle, où nous représentons les territoires,

sur l'importance de ces radios locales associatives implantées dans nos territoires, dans nos quartiers. Elles sont en lien avec tout le tissu associatif, culturel, sportif, institutionnel. Elles sont la voix des territoires. Cette somme

somme qui correspond à une ligne budgétaire d'envoi de lettres aux internautes et au coût des différentes études censées prouver l'efficacité du dispositif. Ainsi, les sanctions prononcées par la Hadopi pour l'année 2021 par l'envoi de lettres seraient suspendues.

D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré en février 2021 contraires à la Constitution les pouvoirs que la loi a donnés à la Hadopi pour identifier les personnes qui partagent les oeuvres sur internet. Quel est l'avis de la commission ? Sur les trois amendements, la commission des finances est réservée. Nous allons demander l'avis du Gouvernement. Pourquoi ? Tous les orateurs ont dit que beaucoup d'efforts avaient déjà été faits par les LFR et par le budget 2021.

Si tel est le cas, je dois reconnaître que je ne vois pas bien pourquoi rajouter 3,5 millions d'euros. Si tel n'est pas le cas, l'avis de la commission évoluera plutôt en faveur de l'amendement à 3,5 millions d'euros,

Bien sûr, comme vous tous, je salue le rôle structurant des radios d'initiative locale, qui jouent un rôle social remarquable sur l'ensemble de nos territoires.

associatives ne sont pas éligibles au dispositif spécifique du fonds de soutien à la diffusion que vous signalez, mais le Gouvernement a souhaité renforcer de manière

pour le calcul des aides versées au titre du FSER en 2021, un assouplissement des critères permettra de tenir compte des circonstances particulières qu'ont subies les radios pendant la crise sanitaire de 2020. Enfin, vous avez voté, dans le cadre de la LFR 4, la création d'un fonds à destination des petites structures de l'économie sociale et solidaire, doté de 30 millions d'euros, et qui sera activé en début d'année prochaine. Je travaille très activement avec la secrétaire d'État Olivia Gregoire pour que ce fonds bénéficie aux radios associatives. Vous allez retrouver votre argent, cher Roger Karoutchi, de cette façon. Ces structures font l'objet de toute l'attention du Gouvernement, et je rappelle le rôle fondamental qu'elles jouent en tant que médias de proximité. Les échanges continuent entre les services du ministère de la culture et les représentants du secteur pour mieux accompagner ces structures sur nos territoires. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ces trois amendements. La parole est à M.

ce merveilleux film. Tout simplement, on l'a vu, et notamment pendant la période de crise, ces radios, que l'on ne doit pas considérer comme de la valetaille,

je soutiendrai très volontiers cet amendement.

Il ne faudrait pas, au travers d'une action qui peut apparaître tout à fait légitime, se livrer à un travail de déstabilisation d'une institution tout à fait indispensable. Je souhaite pour ma part

Malet. Cet amendement vise à augmenter le niveau de l'aide au pluralisme des titres ultramarins, car il est impérieux que la presse papier outre-mer ne disparaisse pas. Si cette aide, nouvellement inscrite au projet de loi de finances pour 2021, doit être saluée, madame la ministre, doit cependant consentir un effort financier supplémentaire, au regard de la singularité de la situation de la presse des outre-mer, défavorisée par l'éloignement géographique de ces territoires et par l'exiguïté de son périmètre de vente.

au vu de leur mission de diffusion de l'information locale, régionale, nationale et internationale, sur un territoire où la fracture numérique est prégnante. Quel